La séance est reprise. Mes chers collègues, j'ai été informé que le ministre, un quart d'heure de retard, donc je vais suspendre la séance pour un quart d'heure et sa reprise à 14 heures 45 la séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution européenne sur l'appui de l'Union européenne à la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale en Irak, présenté en application de l'article 73 cas acquiesce du règlement par monsieur Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe, les républicains. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Bruno Retailleau pour le groupe, les républicains pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, chers collègues, en en 2 mots, je voudrais rapidement présenter les raisons de cette proposition de de résolutions, vous en conviendrez, monsieur le Ministre, nous n'en avons pas encore terminé avec Daech et surtout son idéologie mortifère, nous n'en avons pas terminé au Levant ou de semaine en semaine, les attentats se multiplient en Syrie la semaine dernière 16 morts donc, 4 Américains mais aussi en Europe, en France. à Strasbourg. Au coeur. D'une cité au moment d'un marché de Noël, nous n'avons pas terminé avec cette idéologie mortifère. On le voit à de nombreuses reprises et. L'écho funeste de ces crimes abominables résonne encore. Cet écho résonne d'abord sur les anciennes Terres du califat. Il résonne dans le coeur de c'est millions de femmes. D'hommes d'enfants qui ont été suppliciés. D'une façon ou d'une autre, certains sont rescapés, d'autres pas, qu'il soient yézidis, qu'ils soient chrétiens qu'ils soient musulmans Chabaka nous avons dénombré 7, une mission de l'ONU, plus de 200 charniers avec au moins 12000 corps qui reposait danser charniers au moment où je vous parle, mes chers collègues, on dénombre sans doute plus de 3000. Jeune femme yézidie. Qui sont peu détenues comme esclaves sexuelles dans la région, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous sommes ici dans cet hémicycle, et puis il y a la grande cohorte de tous ces déplacés, je parlais de yézidis, ils étaient 550000. 400000 au moins ont été déplacés, les chrétiens, il y a à peine 40 ans était.

non, nous n'en avons pas terminé avec Daech ni avec cette idéologie mortifère parce que désormais, ce qui est devant nous, c'est un immense chantier, le chantier de la reconstruction, reconstruction d'abord politique et à cet égard les élections du 12 mai ont été nouvelle étape dans le processus de stabilisation de l'Irak évidemment, même s'il a fallu plusieurs mois pour former le gouvernement, mais nous connaissons si en Europe des pays, il a fallu quelques mois pour avoir un gouvernement stable signe positif aussi puisque le nouveau gouvernement de Monsieur Adel Abdel Al, a pris un certain nombre d'initiatives et toutes vont dans un sens, là aussi positif pour faire en sorte que l'ensemble des communautés, quelles que soient les origines ethniques et religieuses, puissent se retrouver malgré ces clivages pouvant confessionnel et j'en veux pour preuve d'ailleurs cette décision que le gouvernement irakien a annoncé le 24 décembre de faire de Noël un jour férié, donc cette reconstruction politique même si elle trouvera de nouveaux défis sans doute d'autres obstacles et sur le bon chemin, il y a la reconstruction matérielle et notre pays, et surtout l'Union européenne est en pointe, nous sommes au 1er rang entre 2014 et 2017 c'est pas moins de 650 millions d'euros qui ont été apportées par l'Union européenne et il y a eu une promesse de 400 millions supplémentaires d'ici à 2020, au moment de la du processus de la conférence de reconstruction en février en début d'année passée 2018, je pense que d'autres efforts sont à faire et surtout vis à vis de la corruption, mais cette reconstruction 30, elle aussi, une bonne voie, je pense, Monsieur le Ministre, je pense, mes chers collègues, il n'y a pas de reconstruction matérielle sans une reconstruction immatériel, ce que je veux dire par là c'est que lorsque on voit dans le monde. Ces sociétés qui ont été fracturées par des grandes violences et notamment par des guerres civiles le préalable de toute reconstruction c'est la reconstruction,

qui vont conviction profonde dans la mesure où ce processus permet de stopper le cycle infernal de la violence dans la mesure où pour utiliser les mots d'Arendt ce processus permet d'entrevoir un nouveau commencement, là où tout semblait avoir terminé, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de deux Arendt bien sûr et je mets en garde celles et ceux qui voudraient attendre. Parce que ce serait prendre le risque de la disparition des preuves, ce serait prendre le risque, la disparition des bourreaux ce c'est prendre le risque aussi d'aller un peu d'alimenter ce cycle de la revanche du ressentiment et ce serait finalement préparer. Les dégâts ou de nouvelles guerres civiles pour demain, il nous faut donc réfléchir à faire en sorte que nous puissions aider l'Irak sans ingérence à mettre en place un cadre qui permet à la société irakienne à toutes ses composantes, de se retrouver autour d'une même citoyenneté, je sais que la tâche est difficile et je pense que le cadre doit être spécifique, le cadre d'une justice rendue équitablement. Un cadre spécifique, d'abord parce que la nature des crimes sont très particulier, vraisemblablement un certain nombre d'entre eux, entrent dans les catégories que le droit international a défini depuis Nuremberg, de génocide, de crimes contre l'humanité, la nature des crimes, les auteurs, ce sont pas seulement des Irakiens. Je vous rappelle que plusieurs dizaines des dizaines de nationalités étaient représentées, entre 2014 et et 2017 et puis il y a aussi un contexte particulier et d'une société qui doit se reconstruire effectivement d'une société d'un processus global qui doit permettre à toutes les composantes, encore une fois, de se retrouver dans un même idéal, un idéal irakien, c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette proposition de résolution, c'est la raison pour laquelle je pense que l'Union européenne pourrait prendre un certain nombre d'initiatives, pourquoi l'Union européenne d'abord, parce qu'elle a une légitimité, c'est sans doute la première puissance qui est l'Irak à se reconstruire sur le plan matériel premières légitimité, une autre légitimité, c'est parce que depuis plusieurs années, je pense notamment à la mission Eurojust Irak l'ex-Irak : l'Union européenne s'est engagée dans ce processus pour soutenir un cadre judiciaire qui soit indépendant qui puisse se rapprocher des standards internationaux internationaux et l'Union européenne a adopté il y a en vue un peu moins d'un an une communication ou encore une fois le proposait un appui justement au gouvernement irakien, il s'agirait de proposer ce cadre spécifique, cette justice transitionnelle à dimension internationale qui pourrait voir le jour avec une solution mixte ou des juges irakiens bien sûr pourrait avec des juges internationaux aider ce pays à juger de crimes, encore une fois très spécifique qui n'intéresse pas seulement l'Irak mais qui intéressent la communauté internationale à ce point de de mon exposé dans l'intervention, je voudrais simplement faire une mise en garde et en même temps apporter un éclaircissement il n'est pas pour nous et pour tous les co-signataires de cette résolution, il n'est pas question d'envisager une quelconque ingérence il n'est pas question d'âge, d'imaginer un seul instant que justice pour être rendu à sens de la souveraineté irakienne, je pense que nous visons la reconstruction : nous voulons une réconciliation que penseraient le peuple irakien, si un jour on lui donnait le sentiment que la justice avait été rendue par d'autres évidemment donc cette initiative notre initiative, cette proposition de résolution, ça n'est certainement pas une invitation à une ingérence, ça n'est certainement pas une initiative pour faire en sorte que la justice irakienne viennent sur d'autres brisé que celle qui concerne sa souveraineté simplement et juste un mot, puisque certains d'entre vous pourraient penser mais alors le statut de Rome, la Cour pénale internationale, non, ça n'est pas à nous de juger ça n'est pas nous choisir, c'est du ressort de la souveraineté irakienne de savoir si oui ou non, le pays doit adhérer au statut de Rome pour avoir accès à cette justice internationale et notamment à la Cour pénale internationale, simplement j'observe qu'à plusieurs reprises et notamment avec l'accord de Paris en 2015, l'Irak avait demandé à la communauté internationale, un certain nombre de soutien et d'appui pour l'aider d'ailleurs dans cette justice vis-à-vis des crimes contre l'humanité, donc l'origine de notre initiative collective de cette, de ce projet de résolution, il est là, il n'est pas à rebours de la volonté de de l'Irak, il est au contraire dans un accompagnement et. On a dès des exemples de ces pays fracturé, on a des exemples de Khadr de justice spécifique d'une justice transitionnelle à dimension internationale sans doute que le meilleur, c'est l'exemple du Cambodge, donc je pense que on peut au moins y réfléchir, ce que je veux dire pour terminer très rapidement et pour conclure, c'est que cette proposition, c'est la traduction concrète de la position constante de notre groupe de lésions,

avec une aspiration, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de reconstruction sans Rykiel sans réconciliation, de même qu'il ne saurait y avoir de réconciliation sans justice, je pense, et nous pensons par ailleurs que. Les crimes commis en Irak concerne en 1er lieu les irakiens, l'Irak, mais concerne aussi la communauté internationale, évidemment, puisque nous avons eu un retentissement chez nous en France sanglants de ces crimes et bien sûr je conclus et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président mais, chers collègues, Monsieur le Ministre, je pense qu'il faut que nous pensions à aider l'Irak sans violer évidemment sa souveraineté, tout simplement parce que les victimes de la bas d'ici et de chez nous réclame justice et je pense que nous aurions intérêt là aussi à donner un soutien à l'Irak pour se rapprocher des standards merci de votre attention. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Bruno Retailleau, vient de rappeler l'ampleur terribles, des crimes de masse de l'État islamique, les chiffres de l'épuration religieuse, ethnique qui a connu l'Irak sont terribles : ainsi, en une génération, la population chrétienne d'Irak, a diminué de 75 ce sont 20 siècles d'histoire qui ont été presque balayé en 20 ans, et pourtant il vaste aujourd'hui des populations chrétiennes et membres de minorités religieuses yazidis Chabaks auquel il notamment qui tentent de survivre dans leur pays, en particulier au Kurdistan irakien, une partie des populations qui ont fui l'arrivée de Daech, en particulier dans la région de la plaine de Ninive Aspire à retourner vivre chez elle, d'abord, tout de suite apporter de précisions dont nos débats en commission la semaine d'être passées ont montré l'importance tout d'abord, il ne s'agit pas ici de défendre les chrétiens d'Orient juste parce qu'ils sont chrétiens ni toute autre minorité du fait de son appartenance à une religion ou à une origine plutôt qu'à une autre, il s'agit de tâches et de conserver au Moyen-Orient et à l'Irak, plus spécifiquement pour le texte que Pando discutons aujourd'hui sa véritable identité, l'identité du Moyen-Orient depuis 3 millénaires et d'être un creuset d'époque, des religions et des cultures, cette ouverture, cette capacité à définir un vivre-ensemble qu'il faut sauver et ce pour des raisons morales, bien sûr, mais aussi pour des raisons de sécurité collective il faut la sauver pour des raisons morales, car nous Européens avons appris les cruelles leçons de l'histoire lorsque l'intolérance prend le dessus dans les sociétés et conduit à la persécution de civils désarmés, que ce soit les trop longues guerres de religion en France, la Shoah dans toute l'Europe, ou plus récemment l'épuration ethnique dans les Balkans, l'histoire de l'Europe s'est forgée dans ces épreuves terribles, la mémoire de ces persécutions dont certains sont encore proches nous font nous fait un devoir de nous élever contre ces crimes de masse, que ce soit au Moyen-Orient ou dans toute autre région du monde, mais si certains trouvaient qu'elle ne suffisait pas à ces raisons morales s'ajoutent aussi des considérations très pragmatique de préservation de notre sécurité, les pays dans lesquels on laisse libre cours nettoyé, jeté ethniques et religieux, où les crimes les plus odieux peuvent être perpétrés sans sanction s'enfonce dans une radicalité toujours plus grande, ce qui en fait aussi tout à des menaces pour leurs voisins, or nous savons bien désormais que la déstabilisation du Moyen-Orient, a des conséquences très directe et très concrète sur les pays européens, que ce soit à travers les entreprises terroristes favorisée par la constitution de foyers du en Orient à travers la propagation d'une version fondamentaliste et dévoyée de l'Islam ou par l'émigration, que les troupes de la région provoque par conséquent encourager le maintien chez elle des minorités du Moyen-Orient, c'est agir selon notre conscience mais c'est aussi agir selon nos intérêts, la seconde précision je souhaitais apporter c'est que notre attachement au respect des droits des minorités ne nous fait naturellement pas oublier les innombrables victimes sunnites de l'État islamique, rappelons que cette organisation jihadiste, si elle s'est fixé comme but de persécuter les minorités a plus généralement commis objectif d'éliminer tous ceux qui n'adhère pas son projet criminel, comme le reste de la population irakienne, les sunnites ont aussi été les victimes des djihadistes et l'attention portée à la volonté de détruire des populations entières du fait de leur appartenance religieuse ou ethnique ne nous fait pas oublier les crimes commis contre certains sunnites, je ne m'attendrais pas longtemps sur le contenu de des propositions que Bruno Retailleau, vient de présenter, je rappellerai simplement que s'attachent à la question de la justice transitionnelle c'est-à-dire justice qui permet d'effectuer une transition entre l'état de guerre civile et d'exactions contre et population à l'état de droit, l'idée d'après le traumatisme des crimes commis contre les populations civiles, la société ne peut revenir à un état normal que si les faits justice de ces crimes n'est pas nouvelle, elle était déjà présente dans l'organisation du procès de Nuremberg, on la retrouve ensuite dans plusieurs pays dans lesquels la démocratie remplace la dictature militaire avec des procès des principaux responsables des juntes on en retrouve enfin des versions récentes plus développé, comme par exemple la commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud, mise en place en 1995 pour permettre au pays de tourner la page douloureuse de l'apartheid, tous ces exemples l'illustrent l'importance de la reconnaissance des crimes et la désignation des principaux responsables pour éviter leur occultation et la perpétuation de l'injustice faite aux victimes, en réalité, il ne s'agit pas de régler les comptes du passé et de prévoir une vengeance ou une revanche, mais bien au contraire de permettre les conditions du vivre-ensemble pour l'avenir, il s'agit d'un point important qui explique à la fois l'intérêt que l'Union européenne porte à ce sujet et la proposition de résolution qui nous est soumise la justice transitionnelle vise en même temps le passé, le présent et l'avenir le passé car il s'agit de nommer les crimes pour ce qu'ils sont de les établir de façon claire et précise pour éviter qu'ils ne soient plus tard nier ou contester le présent car il faut permettre au retour chez elle des populations persécutées, or cet objectif déjà ardu sera presque impossible à atteindre, si ces populations ne peuvent avoir confiance dans une forme de justice et être assurés que leurs droits seront reconnu et respecté l'avenir enfin car comment imaginer que l'Irak puisse se reconstruire pacifiquement, s'il n'est pas rendu justice des exactions passées reconnaître les victimes et ce qu'elles ont subi, c'est aussi affirmer leur légitimité de vivre dans leur pays à retrouver leur maison qui ont souvent été détruites ou occupées par d'autres après leur fuite, il faut rappeler également le contexte irakien, qui est celui d'une décrue des combats et d'un début de normalisation politique si l'État islamique n'a pas été éradiqués, il a perdu l'essentiel de son emprise territoriale et ces activistes ont plongé dans la clandestinité dans les zones sous contrôle gouvernemental, c'est aussi ce début de stabilisation qui rend possible d'envisager la mise en place d'une justice transitionnelle, naturellement, nous devons garder à l'esprit de la nature de ce texte, qui n'a pas la force ne m'a normatif d'une loi toutefois cette résolution peut avoir une portée très concrètes, notamment pour guider l'action de l'Union européenne, c'est pourquoi notre commission adopté cette résolution et propose au Sénat de confirmer cette proposition, je vous remercie. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-François Rapin, en remplacement de Monsieur Jean Bizet, rapporteur pour avis de la commission des Affaires européennes pour 5 minutes.

c'est bien modestement bien humblement je remplacerai si tant est qu'ils soient remplaçable président Bizet sur un sujet très grave. Notre commission a adopté le 18 décembre dernier la proposition de lose de résolution européenne sur l'appui européen un mécanisme de justice transitionnelle en Irak déposée par notre collègue Bruno Retailleau et 80 membres du groupe sénatorial de réflexions de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes, le rapport de la commission des Affaires étrangères, va dans le même sens, la défaite militaire de Daech, pas encore définitive d'ailleurs ne doit pas aujourd'hui faire oublier le sort dramatique des communautés chrétiennes et des minorités en Irak. De 860000 en 2014 le nombre de chrétiens est passé à moins de 400000 aujourd'hui, 125000 chrétiens auraient quitté l'Irak pour la seule année 2014, le sort des fidèles des religion syncrétique préislamique n'est guère plus enviable. Le texte que nous examinons aujourd'hui préconise la mise en place en Irak, avec l'appui de l'Union européenne d'un mécanisme de justice transitionnelle à même de faciliter la réconciliation entre les communautés qui composent ce pays, l'Union européenne s'est engagée à de multiples reprises depuis 2003 pour la reconstruction en Irak, notamment au plan financier. C'est dans ce contexte que la proposition de résolution européenne propose le fléchage d'une partie des financements européens vers un mécanisme de justice transitionnelle permettant de qualifier et juger les crimes commis par Daech sur le territoire irakien. Le texte demande en 1er lieu que ce dispositif est une dimension internationale. La proposition de résolution européenne mais judicieusement en avant l'exemple des Chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens, composée de magistrats internationaux et cambodgiens créée afin de traduire en justice les responsables des crimes commis par les Khmers rouges L'Union européenne finance pour partie leur activité, ce dispositif pourrait être dupliqué à l'échelle irakienne, l'ajout d'une dimension internationale doit constituer, en tout état de cause, une des conditions du soutien européen. La proposition de résolution européenne insiste également sur le travail de formation des enquêteurs et des juges. L'Union européenne pourrait renforcer le mandat de l'actuelle mission eux et contribuer à la formation des forces de sécurité irakiennes aux enquêtes sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, une telle option faciliterait indéniablement la coopération avec l'équipe d'enquêteurs des Nations unies chargée de recueillir des preuves en Irak, qui va commencer ses travaux dans les prochaines semaines la proposition appelle en outre à la mise en place d'une mission européenne destinée à former le personnel judiciaire en le sensibilisant particulièrement aux spécificités des instructions visant, crimes de guerre ou Crime contre l'humanité. Une telle mission viendrait compléter tout à la fois le travail des enquêteurs et celui des chambres mixtes que je viens d'évoquer l'Union européenne dispose d'une expertise en la matière, de par le monde, il faut s'appuyer dessus. Je rappellerai pour conclure que l'Union européenne est souvent là pour mettre fin au conflit. Je pense, toutes proportions gardées, à son rôle essentiel dans l'accord du vendredi Saint, qui a fait cesser la guerre civile en Ulster. En Irak, elle peut oeuvrer à la réconciliation des différentes communautés, c'est pourquoi la commission des Affaires européennes, émet un avis favorable sur ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, monsieur le président, Retailleau, nous voici réunis effectivement autour de cette proposition de résolution européenne sur l'appui que pourrait apporter l'Union européenne à la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale en Irak souligner le grand nombre de signataires et le fait que on y retrouve aussi le président, canner le président, Marseille et que, on le voit bien sur l'ensemble des banques, l'ensemble des travées il y a un souci qui ne date pas d'aujourd'hui, on va y revenir depuis plusieurs années sur la terrible épreuve qu'on subit, hé bien un certain nombre de minorités en Irak et au Moyen-Orient, en général, nous sommes en 2019, et je me souviens encore comme si c'était hier, de ce 26 juin 1999 où j'avais eu la chance, je dis la chance à l'époque d'aller à la rencontre de jeunes chrétiens dans une église chaldéenne de Baldi de Bagdad et à l'époque n'est pas l'habitude de voir de jeunes Occidentaux puisque le pays était frappés d'embargo. Le lien était gardé et depuis, hélas, les trajets qu'ils ont fait qu'ils sont conduits illustrant hé bien je crois beaucoup de cas qui effectivement ont touché nous amis nos frères d'Irak. Une famille parti au Canada l'autre venu en France, certains étant resté mais ayant été frappé sur place et donc je crois que nous avons toutes et tous en tête non seulement des vies, des parcours de vie, mais également un certain nombre d'atrocités et tout cela ne peut pas laisser effectivement totalement indemne alors très clairement, aujourd'hui, vous proposez, hé bien de pouvoir donner un certain nombre d'orientations et je vous remercie pour cette mobilisation qui est la vôtre à travers cette proposition de résolution nous partageons totalement votre diagnostic, de paix durable sans réconciliation nationale et il n'y aura pas de réconciliation sans justice cette justice elle est due à l'ensemble des Irakiens victimes de la barbarie djihadiste et tout particulièrement ses minorités religieuses atrocement et systématiquement persécuté par Daech, hein nous pensons en particulier aux chrétiens yazidis et je veux rendre hommage ici au Sénat qui, dès le printemps 2015, à l'initiative des présidents Larché Retailleau a créé un groupe de réflexion rassemblant tous les groupes politiques du Sénat et qui était l'un des premiers à sonner l'alerte sur le drame vécu alors vous évoquiez monsieur Président Retailleau Hannah Arendt et il est vrai que, elle qui a écrit dans Leishman à Jérusalem sur la banalité du mal, on se remet en compte que hélas cette banalité du mal, elle frappe encore et toujours, comment l'inhumain peut se loger. Si facilement dans ce qui est un être humain et face à ces atrocités qui défie l'imagination qui heurte la conscience humaine, je reprends la formule du préambule du statut de Rome de la CPI, il est légitime, nécessaire de pouvoir compter sur une justice à la hauteur qui garantissent qu'il n'y aura ni oubli ni impunité avant de venir au à la résolution présentée aujourd'hui, permettez-moi de revenir également sur les grands fondamentaux de notre engagement aux côtés de l'Irak, parce que depuis 2014, la France se tient aux côtés du gouvernement et du peuple irakien dans sa lutte contre l'organisation terroriste terroriste Daech nous n'avons eu de cesse de mobiliser nos partenaires européens pour l'appuyer dans cette entreprise, aujourd'hui l'Irak se relève l'Irak Aspire à devenir une puissance d'équilibre, capable de tenir à distance les conflits de son environnement régional proche Jean-Yves Le Drian s'est rendu la semaine dernière en Irak et le président comme on était, de ce déplacement, vous avez rencontré les nouvelles autorités fédérales, les autorités du gouvernement régional du Kurdistan et la France a fait savoir justement combien était désireuse de poursuivre son soutien aux efforts de lutte contre le terrorisme de reconstruction et de réconciliation nationale, d'étendre et de densifier le lien forgé dans le combat commun pour construire une paix paix durable, la France a été depuis le début de la guerre contre Daech le 1er soutien des minorités persécutées fidèle à cette histoire qui remonte à François 1er à nos valeurs, aux Liens anciens et étroits qui nous unissent au chrétiens d'Orient mais aussi parce que nous sommes tout simplement convaincu que la diversité religieuse, elle est une part essentielle de l'identité de l'Irak et du Moyen-Orient, et que cette région ne peut pas vivre sans sel, c'est donc une condition de son évolution vers la paix vers la stabilité, la tolérance et la proximité, et je veux d'ailleurs rendre un hommage aussi à l'action déterminée d'un grand nombre d'associations de l'Oeuvre d'Orient également de la credo et confessionnel comme laïc qui se sont engagés en faveur des minorités persécutées du Moyen-Orient alors vous le rappeliez, cette conférence de septembre 2015 conférence de Paris sur les victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient qui a permis d'adopter un véritable plan d'action pour des mesures permettant de créer les conditions d'un retour volontaire sur durable de ces minorités dans leur foyer, cette conférence, nous avons souhaité qu'elle fasse l'objet d'un suivi scrupuleux et c'est ainsi que vos travaux ont été versés au à ceux de la conférence de suivi de Bruxelles en 2018 et que la France en 2000 19 et bien honorera d'accueillir la conférence de suivi, ce sera vraisemblablement au mois d'octobre, et nous y mettrons l'accent sur l'éducation sur l'inclusivité et justement sur la lutte contre l'impunité reviendrai et j'en profite pour émettre le voeu, et bien que nous puissions travailler ensemble à la construction à l'architecture de cette conférence internationale nous avons également fortement soutenu ces communautés sur le terrain, avec ce qu'souhaitaient trouver en France un asile cela bénéficier à plus de 7000 personnes, nous avons mobilisé notre fonds minorité, plus de 20 millions d'euros qui ont permis à une soixantaine de projets humanitaires et de stabilisation, de voir le jour et puis nous sommes particulièrement investi pour permette le retour des chrétiens à Mossoul et dans la plaine de Ninive, l'AFD vient d'ailleurs de lancer un projet de 10 millions d'euros à cet égard Charles Personnaz a été missionné par le président de la République pour proposer une stratégie pour renforcer l'action de la France au Moyen-Orient, dans le domaine du Patrimoine et notre soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région, il a rendu son rapport le 3 janvier naturellement, nous allons nous inspirer très largement pour pouvoir agir, agir encore et toujours une attention toute particulière est portée également à la communauté yézidi, le président de la République s'est engagé auprès de prix Nobel de la paix, Madame Nadia Mourad pour accueillir une centaine de cette femme yézidie, victime de Daech et leur famille en France pour les aider à se reconstruire une vingtaine d'entre elles sont d'ores et déjà arrivé fin décembre avec leurs enfants, nous contribuerons à la reconstruction du site de la même façon, donc très clairement le devenir de ces communautés est une priorité, une priorité que nous mettons en avant naturellement dans notre dialogue bilatéral avec les Irakiens président Cambon a pu le voir la semaine dernière et y prendre part, très directement la France, a plaidé pour très clairement pour que les nouvelles autorités irakiennes face de l'arrêt qu'une conciliation, il l'inclusivité une priorité, nous nous réjouissons que les initiatives pas prise par le nouveau gouvernement est permis par exemple de déclarer Noël comme jour férié, c'est un symbole fort et les symboles sont importants désormais, il faut s'assurer de la mise en place d'une gouvernance inclusive parce que, on le voit, ces minorités, elle revendique d'être tout simplement des citoyens comme les autres et d'avoir également la voix au chapitre. De façon très concrète, pragmatique, puisque la France en 2019 accueillera la conférence de suivi nous ne verrions que des avantages à ce que l'Irak coprésident à nos côtés cette conférence, la lutte contre l'impunité sera un axe fort de cette conférence parce qu'elle était indispensable à la reconstruction de ces communautés de l'ensemble des victimes de Daech et au relèvement de l'Irak et donc naturellement oui nous souscrivons aux objectifs de la résolution qui vous est soumise la demande d'un soutien européen fort à une justice qui soit à la hauteur des crimes commis par Daech en Irak est pleinement légitime alors ensuite vous l'avez dit d'ailleurs président Retailleau il y a le souci des autorités irakiennes hé bien d'agir en exerçant leur pleine souveraineté et vous l'avez dit clairement : pas d'ingérence mais en revanche effectivement le souci de les accompagner, de leur offrir le cadre les moyens leur permettant de mener à bien, hé bien effectivement cette mission et cette tâche de justice dans le respect de leur souveraineté et de leur compétence des milliers de condamnation d'ores et déjà été prononcée contre Des djihadistes mais très clairement, il est important de pouvoir renforcer les capacités de la justice irakienne de l'aider ainsi à lutter effectivement contre l'impunité, nous faisons a-t-il bilatérales avec des programmes de formation des magistrats irakiens en France, nous soutenons également des projets de documentation des crimes commis par Daech notamment à la rencontre des populations yézidis, c'est ainsi que le ministère de l'Europe des Affaires étrangères a financé le récent rapport de la FIDH consacré aux crimes sexuels commis par des jihadistes étrangers contre yézidis hé bien il favorise l'ouverture effective de poursuites judiciaires pour des faits de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, notamment à l'encontre de ceux des djihadistes étrangers qui sont ou seront jugés hors d'Irak nous entretenons un dialogue politique Danse avec l'Irak nous l'encourageons à devenir partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale et intégrer les crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité à sa législation mais nous agissons aussi à travers les Nations Unies en tant que co-parrains de la résolution 23 79 du Conseil de sécurité qui a mis en place cette équipe d'enquête sur les crimes commis par Daech en Irak, appelé unit had cela permet c'est très précieux de recueillir de stocker des preuves de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité pour que la justice puisse passer un jour et puis l'Union européenne, puisque c'est le coeur de la résolution doit évidemment prendre sa part, vous appelez à mobiliser en ce sens, l'action de la mission civile de l'Union européenne, M. Irak son mandat, a d'ores et déjà été élargi à la formation de certains personnels irakiens aux enquêtes sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité évaluons cette formule avant d'envisager une nouvelle extension mais en tous les cas cette piste doit être creusée et puis, nous souhaitons que davantage de fonds européens soient fléchés vers le renforcement des capacités du système juridique irakien, nous le faisons savoir dans les instances européennes et nous le ferons savoir est d'autant plus de force, maintenant une fois que votre assemblée aura délibéré alors vous le voyez mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement partage pleinement votre volonté d'appuyer la lutte contre l'impunité des crimes de Daech nécessaires au relèvement de l'Irak et de mobiliser l'Union européenne en ce sens, le président de la République, inaugurant cette magnifique Exposition à l'Institut du monde arabe, c'était le 25 septembre 2017 disait carapace et nous oblige soyez sûrs de notre engagement pour le présent, c'est exactement sur ces mots que je souhaite terminer en vous indiquant naturellement la sagesse très bienveillante que le gouvernement accorde à cette proposition de résolution. Si merci monsieur le ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Claude au pour la République en marche pour 7 minutes. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des Affaires étrangères de la Défense, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord saluer le travail de sensibilisation et de suivi qu'effectue le groupe de liaison sur la situation des chrétiens et des minorités au Moyen-Orient ainsi que celle des Kurdes, cette proposition de résolution européenne présentée par le président Retailleau et plusieurs de nos collègues préconise établir un Irak un mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale ou mixtes pour juger les crimes commis sur fond de territoire par Daech de 2014 à 2017, elle demande à flécher d'emblée des financements européens pour la création d'une telle dispositif ces dernières années à travers le monde de l'expérience de la justice transitionnelle nous a montré combien cette étape était crucial pour consolider la paix, au sortir d'une période conflictuelle pour rétablir un sentiment de sécurité pour reconstruire un pays et pour réconcilier une nation meurtrie. La justice transitionnelle comprend 4 piliers complémentaires et indissociables, le droit à la vérité avec l'établissement des faits, la recherche des disparus, les archives, le droit à la justice par la création de commissions d'enquête, mais aussi par des actions en justice au niveau national, régional, international ou mixte, le droit à la réparation par exemple par des programmes de réparation individuelle et ou collectives ou des monuments commémoratifs et enfin l'exigence de non-répétition garantis par des réformes institutionnelles, une constitution insuffisamment protectrices des droits de l'homme des institutions de sécurité mais aussi la mise en oeuvre d'un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ces principes-là ont connu sous le nom de piliers Jouannet non du juriste Louis Joinet et pour chacun, de tous les groupes vulnérables, qu'il s'agisse des minorités, des femmes, des enfants de handicapés doivent être spécifiquement protégée pour éviter le retour de discrimination qui ont pu conduire à des conflits. La justice transitionnelle ne se réduit donc pas au droit à la justice et aux mécanismes de justice transitionnelle évoqués par cette PPR en la matière, plusieurs écueils sont à proscrire, premièrement, il faut se garder de croire que ces 4 piliers peuvent intervenir simultanément. Deuxièmement, une précipitation excessive au nom de l'impératif de la réconciliation, tout comme un ajournement permanent sont tous de contre-productif, dès lors, il est plus que souhaitable que le lancement d'un processus de justice transitionnelle implique au préalable que la situation sécuritaire soit entièrement stabilisée, bien sûr, cette nécessité ne doit pas empêcher de commencer à se concerter pendant la phase de stabilisation sur ce qui peut être le rôle et la forme de tels processus. Avec cette me perds et bien que nous souscrivons aux intentions louables portée nous avons toutefois le sentiment d'être long mais dans l'un de ces écueils que je viens d'énoncer, celui de nous trouver dans une précipitation excessive au nom de l'impératif de la réconciliation. En dépit des progrès récents accomplis l'Irak demeure un pays où l'on se déplace encore en véhicules blindés, les forces de sécurité irakiennes appuyées par la coalition internationale contre Daech procèdent encore à des opérations de sécurisation dans le désert, à l'ouest de la province d'Anbar où des combattants de graisse se sont repliés, pour l'heure, la priorité est donc plutôt au retour de la stabilité sécuritaire et de la souveraineté irakienne en combattant la menace terroriste, nos efforts doivent se concentrer sur la situation humanitaire dramatique la reconstruction des bases de l'état des institutions et des services élémentaires assuré par l'État, tout comme la consolidation du fonctionnement légitime des tribunaux de droit commun et la collecte de preuves sur les qui rime perpétré par Daech, préalable indispensable pour la réconciliation nationale. Cela signifie aussi soutenir Bagdad dans la politique inclusive qu'elle mène vis-à-vis de toutes les minorités du pays, la nomination du nouveau 1er ministre Adel Abdel Mehdi en octobre après un compromis trouvé un tous les 2 blocs chiites rivaux qui ont été vainqueur des élections est un signe prometteur. Nous savons par ailleurs que le pays rechigne à se soumettre à la compétence de la Cour pénale internationale. Bagdad n'est pas non plus demandeur d'un tribunal pénal ad hoc international ou mixtes, or le consentement du pays concerné est une condition sine qua non pour la mise en place d'une telle dispositif. Notre prudence est d'autant plus de mise que rien ne nous assure que les Irakiens accepteront de renoncer à l'application de la peine de mort, même dans ce cadre. Aller aussi vite en besogne, empêchant d'emblée un financement européen comprend alors le risque d'être présentée comme une injonction de braquer le pays et d'être contre-productif, les tribunaux mixtes, peut être une solution, mais à condition de s'inscrit dans le cadre d'une souveraineté pleinement recouvré néanmoins une telle modèle Mixa a aussi pu montrer ses limites dans le cas cambodgien où plus de 10 ans ont été nécessaires avant que les chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens ne puisse débuter leurs travaux. Seule une poignée de responsables, a finalement été jugé toute la lumière n'a guère pu être faites, cela a été extrêmement coûteux et la pression exercée sur les procureurs et les juges internationaux comme cambodgien a été telle qu'il a fallu à plusieurs reprises, trouver un remplaçant au démissionnaire. Dès lors, il semble préférable de continuer à défendre la compétence de la CPI et a appelé l'Irak à la reconnaître, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à étudier la possibilité de déférer ces crimes à la CPI d'autant plus que le procureur de la Cour est déjà impliqué dans la collecte des preuves c'est là également, la position de l'Union européenne et celles adoptées dans le plan d'action de Paris dans l'Irak est parti. Notre groupe soutient évidemment le rôle essentiel joué par l'Union européenne à la reconstruction de l'Irak, nous soutenons et croyons la mise en place et la promotion d'un système judiciaire effectif et indépendant irakiens et à la coopération judiciaire, nous partageons l'avis selon lequel les crimes commis par Daech doivent bien sûr être punis. Mais, avec toutes les réserves que je viens d'évoquer le groupe la République préférera s'abstenir. Mais bien sûr avec bienveillance. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion à la parole est à madame Christine Pruneau pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste pour 6 minutes. Monsieur Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, alors cette PPR tente de répondre à 2 questions. Comment s'assurer que la justice soit rendue dans le cas des crimes de masse commis par Daech et comment amorcer dans ce pays, le développement et la paix, l'équilibre est donc fragile la situation en Irak est encore instable, le risque de se retrouver face à une épuration incontrôlée ou à un pardon généralisée existe d'autant plus quand n'adhérent pas au statut de Rome, Bagdad ne pourrait même pas se reposer sur le Tribunal pénal international, alors comment répondre à la demande d'aide du gouvernement irakien, comment gérer la situation ainsi : il serait opportun de maintenir l'aide apportée à l'Irak pour reconstituer ses institutions, notamment judiciaires, nous sommes ici tous d'accord, dans ce cadre, le programme européen lancé en fin 2017 pour aider les forces de police irakienne doit se poursuivre en vue de récolter l'ensemble des éléments d'enquête de la même manière, la mission européenne de renforcement de l'État de droit en Irak doit être relancée, l'accord de partenariat dont nous discutons doit permettre une communication permanente entre Bagdad et les pays européens. Cela est d'autant plus nécessaire au regard des 5000 Européens qui ont rejoint Daech en Syrie ou en Irak de 2011 à 2016, à ce titre, le plan d'action de Paris présenté en 2015 doit être pleinement mobilisés ensuite comment conforter la reconstruction d'un pays ne doit pas forcément signifier sa mise sous tutelle la volonté exprimée par les autorités irakiennes de pouvoir juger sur son sol Les actes qui relèvent de sa législation doit être écouté, monsieur le Président Retailleau, vous l'avez précisé au niveau de la non ingérence que penser alors de cette proposition de résolution la volonté de créer un mécanisme judiciaire proche des C. E. T. qui était rappelé par mon collègue précédents trou tentent de trouver un équilibre subtil mais sans pourtant y arriver pleinement, il est vrai que l'absence de reconnaissance des crimes contre l'humanité dans la loi antiterroriste irakienne de 2014 pose un problème majeur, il est vrai aussi que l'ONU pointe depuis plusieurs années, le risque que les juridictions nationales irakiennes se montrent peu enclines à juger les crimes commis par Daech toutefois, rappelons-nous les limites importantes, des soutes, c'est, je pense notamment à la langue lenteur extrême des procédures et au final au jugement d'appel 10 anciens responsables Khmers en 20 ans de plus dessaisir Bagdad d'une partie de ses prérogatives judiciaires pourraient ralentir considérablement sa reconstruction sociétale et institutionnelle ne sous-estimons pas l'importance du travail judiciaire dans Le Devoir de mémoire d'un État. Comme le pointe la résolution l'Irak et tout finale un État composite où ont cohabité musulmans, chrétiens Chabaks qui hésite et autres, comme nous l'avons tous précisé la demande légitime des autorités irakiennes de pouvoir juger sur son sol les criminels ou disons plutôt les terroristes islamistes et leurs complices pourrait pleinement participer à la reconstruction de l'Irak en Aquitaine, en incluant l'ensemble des irakiennes et des Irakiens et c'est sur cette notion ensemble des Irakiens et des Irakiens que j'émets quelques réserves par rapport à l'écriture de l'alinéa 7 qui propose spécifiquement qui note spécifiquement, d'une part les victimes chrétiennes et d'autre part, les victimes venant d'autres minorités religieuses cette distinction dans le texte me semble alors que votre intervention, monsieur le Président Retailleau sur ces points préciser dans votre intervention, vous avez absolument mélanger toutes les religions, mais ça ne correspond pas au texte sur lequel j'interviens car pour nous, vous comprenez la nuance, j'espère, une victime de Crime de masse de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité reste une victime, quel que soit, Régine, sa race, sa religion, toutes les victimes doivent avoir les mêmes droits. Donc si vous voulez, notre groupe a donc sur ses réserves là vraiment sûrement seulement sur ses réserves, nous allons nous abstenir avec une certaine bienveillance en fait parce que nous notons quand même, elle prône un renforcement de la coopération en respectant la souveraineté de l'Irak, je vous remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Yannick Vaugrenard, pour le groupe socialiste républicain pour 10 minutes. Monsieur le ministre. Messieurs les rapporteurs, monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le président de la commission un une mi-après la fin des combats contre l'État islamique en Irak, le pays a donc entamé un long travail de reconstruction, 4 années de guerre ont en effet non seulement partiellement détruit le pays mais aussi fait des milliers de morts, bien sûr, c'est l'ensemble du peuple irakien, qui est concerné, mais n'oublions surtout pas que Daech avait ciblé un certain nombre de communautés. à ce titre, bien sûr, les chrétiens d'Orient ont eu à subir, nous ne savons de très lourds, massacre les pires exactions accompagnée dans ce triste bilan parlait yézidis les Turkmènes les Kurdes ou encore les shabbat, il convient aussi de souligner dans ces horreurs que le terrorisme de l'État islamique a aussi ciblé et durement le monde musulman. à l'heure actuelle, les survivants recherche toujours leurs disparus, des milliers de corps sont enfuis sont enfouis dans les ruines des villes où ont été jetés dans des charniers. Ce sont, aujourd'hui, pour être précis, 202 de ces charniers de l'État islamique qui ont été découverts ou soeur ensevelies entre 6000 et 12000 corps, beaucoup reste encore à faire pour les familles et leurs victimes, la France joue pleinement son rôle, vous l'avez rappelé monsieur le ministre, depuis 2014, son rôle de soutien auprès de l'Irak pour sa reconstruction, chacun a noté la présence du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, voici quelques jours à Nadjaf, la ville sainte du sud du pays où les pèlerins chiites du monde entier viennent se recueillir sa rencontre avec l'une des plus hautes autorités chiites d'Irak, fut l'occasion d'annoncer un nouveau prêt d'un milliard d'euros sur 4 ans pour des projets de reconstruction, il vient compléter un 1er prêt de 430 millions accordés en 2017 l'absence et la déliquescence des services publics, principalement les coupures d'électricité, rendent la vie quotidienne, particulièrement difficile pour les Irakiens, au-delà des mots et des déclarations d'intention, nous pouvons, je pense que nous féliciter de l'investissement congrès concret de la France auprès de notre partenaire historique j'en viens au texte qui nous est présenté aujourd'hui la proposition de résolution demandant donc l'appui de l'Union européenne à la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale en Irak, je voudrais tout d'abord donné les raisons pour lesquelles nous sommes favorables à cette proposition de résolution, la 1ère c'est d'exprimer notre détermination à lutter absolument contre toute impunité, c'est un impératif, à la fois moral, juridique et politique, le droit à la vérité, le droit à la justice le droit à la réparation et finalement probablement la meilleure garantie de la non-répétition la 2ème raison, c'est que l'Europe venait montrer son exigence humaniste, si elle est déjà à la reconstruction de l'Irak, parallèlement, elle doit aussi soutenir la mise en place d'une justice transitionnelle de son moi sont indissociables et non pas à se succéder, bref en termes d'exigence humanitaire, il n'est jamais urgent d'attendre, d'autant que dans le cas de l'Irak et du Moyen-Orient, en général, notre pays a une responsabilité historique particulière, toutefois, celle-ci doit passer autant que faire se peut, par une décision européenne au-delà l'aspect pratique et juridique, un engagement de l'Europe en faveur d'une justice transitionnelle en Irak, a une valeur symbolique forte, c'est une question essentielle au nom du respect des droits de l'homme, mais c'est peut-être aussi finalement un gage de sécurité future pour notre propre continent. La France parce qu'elle fut durement touchés par l'État islamique est dans son rôle lorsqu'elle souhaite pousser l'Union européenne à prendre sa place et ses responsabilités dans ce domaine avant de, poursuit mon propos mais collègue je voudrais ici, rendre hommage à ceux qui, par la force de leur engagement, par la force de leur détermination et trop souvent. Par le sacrifice de leur vie auront permis de faire reculer Daech même si l'État islamique n'est pas totalement éradiquée, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous pouvons précisément : imaginez une autre étape d'évolution vers la démocratie, qu'il soit chaleureusement remerciés pour leur engagement cette seconde étape indispensable, hé bien nous y sommes et l'histoire nous enseigne depuis toujours face à la nature totalitaire et génocidaires la réponse uniquement militaire ne suffisent, mais la reconstruction est certes une étape essentielle, mais elle doit être accompagnée de la volonté de combattre le totalitarisme, par la force du droit et de la justice qui doivent succéder à la force militaire, la paix ne se gagne pas seulement avec les armes, elle se gagne aussi par la puissance des valeurs de respect mutuel, de tolérance et d'acceptation des différences sur lesquels doivent reposer la justice et le droit, c'est la raison pour laquelle il est indispensable de solder les horreurs passées sans pour autant à l'évidence les oublier pour cela la non-impunité des crimes est une ardente obligation est un passage obligé, sans quoi aucune réconciliation n'est envisageable, aucune réconciliation n'est possible chez Lu but même profond d'un mécanisme de justice transitionnelle, la France, je l'ai dit, doit prendre sa place, l'Europe, tout autant, ainsi que la communauté internationale, à l'évidence, c'est pourquoi je voudrais également vous faire peur, monsieur collègue de ma conviction profonde, le soutien européen re mécanisme de justice transitionnelle devra prévoir que celui-ci est forcément une dimension internationale, il faut qu'ils soient associés magistrats irakiens et magistrats internationaux en vue notamment de mieux prendre en compte le droit international et les incriminations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, à cet égard, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, je mets je prendre également l'exemple cambodgien le processus vérité a pour ce pays finalement bien fonctionné, l'association des juges cambodgiens et de juges étrangers a permis à ce tribunal de faire sereinement son travail et aux victimes d'être reconnues comme telles, c'est en effet la reconnaissance des crimes qui peut aider à entrer dans un processus de réconciliation et faciliter le chemin de démocratisation pour ensuite permettre une justice véritablement indépendante des autres pouvoirs, je ne nie pas tout ce qui reste à parcourir pour aboutir à la mise en oeuvre d'mécanismes le contexte régional ne facilitera pas cette démarche comme les jeux de dupes ici joue, c'est pourquoi l'Europe doit être volontariste tout obstacle mérite d'être surmonté l'Europe, de par son histoire, de par ce qu'elle a traversés et a su surmonter est une voie particulière à part et à ce titre, il se trouve que les parfois respecter l'enjeu est important : il s'agit aussi d'exprimer la capacité de l'Union européenne a projeté en quelque sorte des valeurs humanistes fondamentales et de respect des droits de l'homme au nom desquels les crimes ne peuvent rester impunis, il l'envoie à la fois de notre crédibilité, mais peut-être aussi de notre sécurité présentes et futures, actuellement nous donnons le sentiment parfois au niveau européen, d'être paralysé par des Jeux régionaux qui mène, Turquie, Syrie, Iran et Russie, de plus, l'imprévisibilité de la politique américaine et le fait que le soutien américain n'est plus indéfectible ont et vont à l'avenir, profondément bouleversé nos stratégies européennes habituel. Pour autant, mais, chers collègues, nous ne pouvons nous permettre aucune frilosité, l'Europe est plus que jamais face à ses responsabilités, elle a trop souffert de crimes contre l'humanité pour en négliger sa condamnation partout ailleurs dans le monde, il est donc urgent d'agir et fondamental de procéder à la reconstruction de l'Irak, mais cela ne doit pas empêcher d'aborder dans le même temps, les questions juridiques et de droit international dans l'un ne va pas sans l'autre, je le redis, pour finir, l'Union européenne doit affirmer avec détermination sa volonté de lutter contre toute impunité pour des raisons d'ordre moral, politique et juridique, elle doit défendre avec force son exigence humaniste et prendre toute sa place et ses responsabilités, la communauté internationale et l'ONU doivent prendre la leur aujourd'hui, mais son collègue, prenons les nôtres pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de cette proposition de résolution. Merci, cher collègue, dans la suite de la distance. C'est en général la parole est à monsieur Olivier Léonard pour le groupe RDSE pour 6 minutes.

Monsieur le président. Monsieur le président de la commission, messieurs et mesdames les rapporteurs, seul le ministre, chers collègues, la paix en Irak repose non seulement sur sa reconstruction matérielle. Et politique, mais aussi sur sa reconstruction morale. Qui devra évidemment passer par la réparation des exactions commises depuis 2014 par Daech contre la population civile, c'est le sens de la proposition de résolution qui est soumise aujourd'hui à notre examen, la nature, l'ampleur des crimes recensés en Irak, justifie que l'on encourage tous les outils qui iront dans le sens d'une politique de réconciliation entre toutes les communautés vivant sur le territoire irakien. j'ai besoin de rappeler ici l'horreur des actes perpétrés par les djihadistes de rappeler les meurtres, les tortures, les déplacements forcés, les viols et la réduction d'en esclavage des milliers d'hommes et de femmes, doit-on rappeler l'enfer vécu par les minorités chrétiennes par le yézidis par les minorités kurdes et en général l'enfer vécu par tous les musulmans qui n'adhéraient pas au califat, doit-on rappeler que certaines de ces exactions relève, disons-le clairement du Crime contre l'humanité. C'est pourquoi la réponse judiciaire doit être à la hauteur des drames vécus à l'instar de ce qui a pu être fait par exemple Pour l'Afrique du Sud, ou pour le Cambodge, nous savons que ces grands moments de vérité judiciaire permettent à la fois de satisfaire les attentes individuelles mais également de refonder une mémoire collective apaisée par le sceau de la justice, une étape nécessaire au retour à l'apaisement et à la paix dans ce cette perspective et sachant que l'Irak ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, il me semble qu'un mécanisme de juridiction de justice transitionnelle à dimension internationale et l'une des réponses que l'on peut apporter aux victimes comme nos collègues rapporteur l'ont rappelé, c'est une initiative qui recueille l'assentiment de l'Union européenne bien sûr, je pense que la réussite d'untel, dispositif est conditionnée au minimum par le respect de 3 principes. Transparence capacité l'outil j'judiciaire irakien et bien entendu l'adhésion sincère déshérités des autorités irakiennes à une entreprise de réconciliation s'agissant de la transparence, l'accueil par l'Irak depuis 2017, une équipe internationale d'enquêteurs au titre de la résolution 23 79 du Conseil de sécurité des Nations unies est plutôt un bon indicateur. En ce qui concerne la capacité de l'outil j'du judiciaire, la proposition de résolution avance 2 pistes, le lancement d'une nouvelle mission d'assistance européenne dans le domaine judiciaire afin de former des magistrats, ainsi que l'élargissement de la mission EUTM EUTM Irak afin d'y intégrer la formation aux enquêtes sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, je soutiens, bien que ce soutien, bien évidemment, ces orientations, même si je sais que tout cela demandera du temps et, s'agissant en particulier de la seconde piste, elle risque de s'heurtée au fait que la loi antiterroriste irakienne ne prennent pas en compte la notion de Crime contre l'humanité. S'agissant enfin l'état d'esprit du pouvoir en place. On peut aussi entre optimisme et pessimisme car on le sait bien, les autorités actuelles sont soucieuses du respect de leur souveraineté et par conséquent les missions régaliennes qui lui sont attachés. Alors l'adoption de cette proposition de résolution constitue un encouragement au lancement d'un processus de réparation qui est due à tous ceux qui ont souffert des atrocités exercée par Daech. Ce sera également un signal positif pour favoriser plus rapidement le retour des personnes réfugiées ou déplacées. En attendant, la communauté internationale doit demeurer vigilante. Car le bon rétablissement des États, des institutions et des principes d'une justice démocratique en Irak, des bancs dépend fortement des contours de la paix dans toute la région et à cet égard, personne n'ignore que la situation est encore bien fragile, que ce soit en Syrie ou en Irak, la reconquête des territoires ne signifie pas la fin du terrorisme islamiste, alors oui. Nous devons soutenir tous ceux, toutes celles et ceux qui ont été et qui seront, et qui sont encore aujourd'hui. Nos meilleurs alliés contre Daech je pense évidemment aux Kurdes le peuple kurde qui s'est battu en première ligne sur tous les fronts et qui a remporté de grandes victoires contre le terrorisme islamique en Irak comme en Syrie, alors oui si nous en sommes là aujourd'hui, c'est surtout grâce à eux il faut jamais l'oublier en 2 en début de l'année dernière lors des attaques menées par le gouvernement turque à Afrine j'avais déjà fait part de mon indignation et à cette époque, les troupes américaines étaient encore présentes et la Turquie devait forcément en tenir compte mais que va-t-il se passer demain lors du retrait des troupes américaines dans cette région en Syrie l'Euro Java et non Par et on ne peut pas exclure une offensive de Damas, qui ne reconnaît pas les forces démocratiques syriennes comme légitime et au sein de laquelle je le rappelle, se trouvent de nombreux Kurdes vous l'Euro compris, vous l'aurez compris le peuple kurde est gravement menacée mis en étau entre la Syrie et la Turquie et le président Macron a eu raison de de d'appeler la Russie à préserver les Kurdes, chers collègues, si nous voulons encourager une peur du rapport Charpin dans cette région du monde, nous ne pourrons pas le faire en tournant le dos au peuple kurde, la communauté internationale de doit pas faire preuve d'amnésie, elle ne doit pas oublier ses alliés, elle ne doit pas abandonner celles et ceux qui ont combattu victorieusement contre les djihadistes, que ce soit Arakawa Kobané j'ajouterai que les Kurdes continuent qui constitue aujourd'hui à lutter, continuer

dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Louis Masson pour le groupe des non-inscrits pour 3 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, il est évident que comme tout le monde je suis horrifié par les exactions de l'État islamique et par tout ce qui se passe comme pratique de scandaleuse par rapport au droit de l'humanité dans les pays arabes, ceci étant en France en particulier, c'est quand même facile de se donner bonne conscience. Il y a des centaines de milliers de morts en Libye. Des centaines de milliers de morts en Syrie. Mais la faute à qui. Tu sais qui a été enclenchée, la guerre en Libye pour déstabiliser le gouvernement de Kadhafi qui n'était pas un ange, je suis tout à fait d'accord que Monsieur Kadhafi n'était pas un ange, mais du temps de Kadhafi il y avait peut-être 1000 ou 2 1000 morts par an, depuis que la France est allé faire la guerre chez Kadhafi et c'était Monsieur Sarkozy. Qui pour des raisons éventuelles d'intérêt national et peut-être pour d'autres raisons moins avouables chez Monsieur Sarkozy qui a été faire bombarder par les avions français du colonel fin de monsieur Kadhafi qui essayaient de se restructurer, hé bien, bon, la France est fière, on a renversé Kadhafi et au lieu d'avoir quelques milliers de morts par an, on a 100000 bon en Syrie, Monsieur Hollande a voulu renverser le gouvernement Assad monsieur Hollande a fait tout ce qu'il a pu, il était à la pointe du combat, on a rouvert, on a essayé de renverser Assad hé bien du temps d'Assad, il y avait un certain nombre de milliers de morts actuellement, hein, les morts se comptent par centaines de milliers, hé bien nous, Français, nous n'avons pas à être fiers de nos gouvernements successifs tout comme nous n'avons pas à être fiers de la politique que conduit Monsieur Sarkozy actuellement au Yémen, sait qu'on Yémen : il y a tout le monde sait qu'au Yémen, il y a des crimes de guerre et des crimes de l'humanité commis par l'Arabie Saoudite, bon hé bien l'Arabie Saoudite ces cachotteries mais on leur tire le tapis rouge, alors il y a 2 poids, 2 mesures, on n'admet pas que Monsieur Assad trash si telle ou telle chose, mais le roi d'Arabie, alors lui il est sacré, il fait ce qu'il veut, il assassine les gens il vont bombarder les populations civiles au Yémen, il fut un génocide contre et on lui dit merci et en plus on le vend les armes nous vendons actuellement à l'Arabie Saoudite, les armes qui Servent à commettre des crimes de guerre, oui Monsieur le Président, ce qui veut dire que nous avons du sang sur les mains, par la faute de certains de nos dirigeants, que ce soit en Libye vis-à-vis de la Libye vit la résolution vis-à-vis du Yémen, votre avis : je crois que c'est scandaleux à ce niveau-là, merci Monsieur le Président, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je vous je vous quitte, je je vous bloque pas. Merci, merci, cher collègue. Non à la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Marie Bockel pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Merci la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui résulte du travail oui de notre groupe de liaison, nous sommes nombreux sur tous les bancs en faire partie et de l'engagement constant de son président, Bruno Retailleau, ce mécanisme de justice transitionnelle qu'elle promeut est nécessaire pour éviter la vengeance ou de suite aux horreurs commises par Daech et permettant la reconstruction du pays, en tout cas y contribuer que la réconciliation des communautés s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de celle votée par notre assemblée, le 6 décembre 2016 et qui a invité le gouvernement à l'époque à utiliser toutes les voies de droit pour reconnaître les crimes de génocide et crimes contre l'humanité, les crimes de guerre perpétrés contre les minorités ethniques et religieuses et les populations civiles en Syrie et en Irak, les intentions de la présente proposition de résolution sont donc profondément bonne cependant, cela ne suffit pas, encore faut-il qu'elle se traduise en actes, car comme le dit fort bien : Pierre de Villiers gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix, la présence des chrétiens au Moyen-Orient et bien antérieure à l'arrivée de l'Islam, ce sont les descendants des premières communautés chrétiennes et ils sont partie intégrante de l'identité de la région de plus, il ne faut pas oublier que la France entretient une relation historique d'amitié avec ces communautés qui découle de l'accord dit des décape, utilisation de 1536 le pape Jean-Paul II considéré, lui, que la situation des chrétiens dans leur pays est révélatrice de l'ensemble du pays, plusieurs collègues l'ont dit, ça n'est pas que la question si sensible des chrétiens et des minorités, c'est la question du devenir de ces pays, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui et si, au début du 20ème siècle, un habitant du Moyen-Orient sur 4 était chrétien, il ne représentent désormais plus que 3 pourcent comme vous le savez, les chrétiens irakiens perçus comme des alliés de l'Occident, ont vu leur situation se dégrader considérablement ces dernières années, il en va de même pour plusieurs religion syncrétique et particulièrement yézidis qui rassemble des centaines de milliers de personnes l'émigration de toutes ces minorités s'est accélérée massivement de par la stratégie Daech visant à supprimer systématiquement toutes les formes de diversité culturelle et religieuse, cela a été dit, la moitié sont partis en Europe outre-Atlantique et nous reviendrons pour la plupart jamais quant à l'autre moitié, elle s'est réfugiée dans les pays de la région essentiellement limitrophes et pour beaucoup aspirent à retourner dans leur pays et verront aussi que nous devons tendre la main car, comme l'affirmait la militante yézidie, Prix Nobel de la paix Nadia Mourad lors de son passage à Paris, le 22 décembre dernier la priorité pour les il dit et de récupérer leurs Terres, ce qui passe d'ailleurs par la reconstruction également de cette région, par ailleurs, je suis convaincu qu'aider les minorités à rester en Orient, nous sommes convaincus, je crois, tous contribuent à consolider un front contre l'extrémisme je tiens également à souligner que cette proposition de résolution trouve un écho particulier au regard de l'annonce le mois dernier du retrait programmé des forces américaines en Syrie, en effet, cela donne un rôle crucial à l'Irak comme base arrière dans la lutte contre Daech car la guerre contre l'arrêt je n'est pas terminé en Syrie, beaucoup l'ont dit, c'est pourquoi quelque 350 militaires français, monsieur le ministre reste déployée en Irak pour lutter contre les derniers combattants de l'État islamique et la France continuera en tout cas c'est notre attente forte à soutenir les Kurdes dans cette lutte, tend donc à redevenir un acteur diplomatique majeur sur la scène régionale, nous avons d'ailleurs pu observer une minute si y a fait allusion, le ballet diplomatique jouer à Bagdad la semaine dernière avec, côté français, la visite de notre ministre d'affaires s'étrangère cette visite, je crois, s'inscrit dans la continuité d'un engagement constant de la France aux côtés du peuple et du gouvernement irakien pour la mise en Inde, une politique de réconciliation nationale et pour reconstruire le pays dans ce domaine-là, en tout cas, nous avons été, gouvernement après gouvernement constant cet engagement s'est traduit par un soutien politique, diplomatique, militaire et humanitaire, cet engagement de la France tant d'autant plus à se consolider que de réels progrès ont été constatés ces dernières mois, ces derniers mois, vers une politique inclusif, comme l'on dit vis-à-vis de toutes les minorités du pays ce dont peu ce dont on ne peut que se réjouir, la prévention de l'émergence du djihadisme passe également par le construction et économique de l'Irak et c'est pourquoi je salue aussi l'annonce la semaine dernière d'un prêt de la France d'un milliard d'euros sur 4 ans à Bagdad. L'Union européenne, quant à elle, s'est fortement impliquée depuis le début, depuis le début de la 2ème guerre dès 2003 pour soutenir les efforts de reconstruction de l'Irak, l'enjeu de l'Union européenne aujourd'hui consiste en particulier à soutenir le gouvernement irakien pour pour mettre en oeuvre une réforme de la justice et a procédé à un alignement du droit irakien sur certains standards internationaux volontairement, comme l'a dit en introduction, tout à l'heure, le président Retailleau mais tout de même c'est important en intégrant notamment les incriminations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui rejoint d'ailleurs sous une forme plus aboutie, la proposition de résolution de notre collègue Nathalie Goulet sur la création d'un tribunal pénal international chargé de juger les djihadistes européens ayant servi sous Daech ou avec Daech, la mise en place d'une justice transactionnelle en Irak à dimension internationale est essentielle afin que ce pays puisse panser ses plaies se reconstruire la France doit donc à son niveau, veiller à ce qu'une partie des financements européens à destination de l'Irak soit dédié à la concrétisation effective de ce mécanisme car, par-delà, de l'Irak, il en va ainsi de la stabilité de toute une région quand je disais il y a l'intention, la résolution il a. Il y a les actes l'amour et les preuves d'amour là, forcément, il y aura des arbitrages, y compris dans les discussions sur l'affectation des fonds européens et c'est vrai que je l'évoquais moi-même tout à l'heure, la dimension de reconstruction économique est essentiel, bien sûr, mais il ne faut pas que sur ce plan il in fine est une sorte de comme souvent de variable d'ajustement, alors que c'est un domaine où avec des moyens assez limités, on peut faire un travail considérable et cette dimension humaine psychologique, politique de réconciliation, d'ailleurs tous les, tous les après-guerre dans notre humanité D. récentes décennies montre que ces moments de construction d'une réconciliation, y compris sur d'autres continents sont des moments essentiels pour la suite, pour la paix à venir à consolider ou pour les risques de conflits nouveaux qui peuvent resurgir à tout moment, donc c'est au fond encore beaucoup plus important. Qu'il n'y paraît, par rapport à tous les enjeux de ce pays qui a tant souffert mais la problématique de la justice transitionnelle en Irak s'inscrit également dans le cas du large, de la lutte contre le terrorisme de ses effets résiduels, avec notamment l'enjeu des revenants ces djihadistes originaires de l'Union européenne, outre le fait qu'il est essentiel pour les victimes de voir juger les combattant Daech là où ils ont commis leur acte, mais aussi l'Europe en même temps a d'autant plus intérêt à soutenir la justice irakienne que cela sert sa propre protection pour toutes ces raisons, le groupe Union centriste votera lui aussi cette proposition de résolution, je vous remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion. Non, la parole est à monsieur Joël Diario pour le groupe, les indépendants pour eux 6 minutes. minutes. Ce président c'est le Ministre, monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, mais sa collègue, je tiens à saluer, au nom de mon groupe, cette résolution du Groupe de liaison de réflexions de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes, si l'Irak est reconnue comme un État de droit souverain par ses partenaires internationaux de nombreuses insuffisances sont constatés, la peine de mort et pratiquer des conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies, la notion de Crime contre l'humanité n'existe pas dans la législation irakienne la Cour pénale internationale n'y est pas reconnu. les criminels se nourrissent donc d'un sentiment d'impunité, quelles que soient les fêtes qu'ils ont commis, or les poursuites pour crimes contre l'humanité sont primordiales du point de vue des victimes civiles, c'est la seule manière de faire en sorte que ces victimes soit entendu et surtout qu'elle puisse obtenir justice et parmi ces victimes, ça l'intéresse, a été rappelé par le président Retailleau il ne faut pas oublier les chrétiens d'Orient qui ont souffert de nombreuses exactions en Irak au cours des 3 dernières décennies environ 80 pourcent de ces chrétiens ont dû quitter le pays et comme ça a été dit, alors que c'était 1,2 millions dans dans les années 80, ils ne sont plus aujourd'hui que 300000 ils sont délaissées par le gouvernement irakien et terrifié par un avenir incertain. Traditionnellement, au nom de la recherche de la réconciliation nationale, l'approche dominante reposait sur une PAC un pacte de l'oubli, fondée sur l'amnistie et l'amnésie, autrement dit sur l'oubli juridique et l'oubli social autres temps autres moeurs cette vision d'une amnistie amnésie cicatrisant les plaies n'est plus admissible aujourd'hui la recherche de la vérité s'impose progressivement comme une partie incontournable des droits de l'homme aujourd'hui les mécanismes de justice transitionnelle se compose de poursuite en justice des auteurs de crimes, de la mise en place d'initiatives en faveur de la recherche de la vérité de l'octroi de réparation aux victimes de violations de droits de l'homme et de la réforme des institutions judiciaires et politiques pour éviter la répétition de telles violations, il est nécessaire de regarder ces mécanismes comme un ensemble indivisible. Il y a une relation d'interdépendance de complémentarité entre par exemple l'réparation et révélation de la vérité, pour être efficace, une mesure ne serait opéré isolé ment et à l'écart des autres, la réconciliation décrit un état dans lequel les relations sociales sont caractérisés par une sorte de confiance civique est basée sur le respect, ce que nous, Occidentaux pourrions schématiquement résumée par notre savoir-vivre ensemble. Des mesures de justice transitionnelle peuvent contribuer à édifier des institutions dignes de confiance, réconcilier les victimes et leurs bourreaux, assurer la primauté du droit à panser les plaies du passé et rétablir une culture basée sur le respect des droits de l'homme, elles permettent de rétablir des relations sociales fondées sur la confiance civique ancrée sur le respect pour rétablir à certains vivre-ensemble aussi la justice transitionnelle n'est pas simplement une justice rétrospectives, mais aussi de justice prospective, on ne cherche pas seulement à réparer les événements passés, mais surtout à unifier une nation sur des bases différentes, plus juste, il s'agit de restaurer une société qui a été brisée par un conflit et l'accompagner vers l'harmonie et la paix, la situation irakienne depuis 25 ans démontre combien la transition démocratique et institutionnel est importante, la mise en place de ce mécanisme donc souhaitables, il s'inscrit plus largement dans la continuité des actions déjà menées par l'Union européenne et par les nations une vue ni pour aider ce pays à se reconstruire un système judiciaire indépendant de vendre des comptes est indispensable pour permettre à ce pays d'aller de l'avant de se reconstituer et surtout de réconcilier ces communautés. On peut regretter que les orientations fixées par le Conseil de l'Union européenne en janvier 2018 concernant la justice transitionnelle en Irak et en Syrie n'est pas précisée, malgré ce que ce sujet soit un des axes forts prévus tout le contexte et sa maison neuve pour relever les 6 défis identifiés dans la stratégie de l'Union européenne, cette initiative doit être appuyé est rendu concrète en insistant notamment sur la sensibilisation à la formation des juges et en s'assurant que les fonds nécessaires soient débloqués. Sans tomber dans la gérance et en veillant à ne pas heurter la souveraineté de l'Irak et de s'et sa sensibilité, il convient d'avoir un regard attentif aux procédures mises en place et apporter conseil et expertise par le biais d'une assistance judiciaire afin d'insuffler dans le droit irakien les principes juridiques de droit international standards qui initie figurent pas, il faut aussi être en capacité de vérifier que toutes les communautés ayant été affectés soient traités de la même manière, y compris les djihadistes français le groupe les indépendants républiques et territoires approuve donc la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale en Irak comme une étape indispensable pour permettre aux familles des victimes de faire leur deuil et en obtenant, reconnaissance et réparation justice doit être rendue pour permettre la réconciliation entre les communautés en Irak, c'est un des piliers de la reconstruction politique de ce pays, merci. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 1979 Simone Veil, première présidente du Parlement européen, disait que l'Europe était le grand dessein du 21ème siècle et qu'elle devrait faire entendre sa voix et défendre des valeurs la proposition de résolution européenne de Bruno Retailleau, s'inscrit parfaitement dans ce grand dessein et je voudrais le remercier très sincèrement d'avoir pris cette initiative, tout comme celle de la création, en 2015, d'un groupe de réflexion sur les chrétiens et les minorités d'Orient, la France et l'Europe, patrie des droits de l'homme est garante de paix ne pouvait rester immobile face aux crimes barbares de Daech et de sa vision du monde fondée sur le déni de l'égale valeur et de l'égale dignité de toute vie humaine ainsi que sur l'élimination de tous ceux qui s'y refusent les crimes les plus graves qu'soient génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ont été commis entre envers les minorités, c'est ethniques et religieuses chrétiens yézidis mais aussi chiites, kurdes, turkmènes demander Saber hein ou encore Chabaks, tous ont été victimes d'exactions d'une indicible cruauté, ils ont été spoliés convertis de force battu enlever, violer, torturer, mutiler réduire en esclavage, notamment sexuels ou massacrer leurs lieux de culte vandalisés ou détruit, c'est une épuration permanente et systématique, un projet de nature génocidaire qui a été mis en oeuvre au coeur du Croissant fertile, berceau de tant de peuples de civilisation et de religions qui ont façonné l'histoire humaine, ce sont des identités multiséculaire que Daech a tenté de faire disparaître avec un certain succès puisqu'ils ne sont plus que 300000 chrétiens dans cette région, ces crimes ne peuvent rester impunis après la réponse des armes, nous devons poursuivre notre combat contre l'ogre barbares sur le terrain des valeurs du droit et de la justice dès juillet 2014 j'avais initié en appel parlementaire signée par plus d'une soixantaine de collègues pour demander à la France d'appeler le Conseil de sécurité de l'ONU à saisir la Cour pénale internationale sur les crimes de Daech en vain un an plus tard, après avoir constaté moi-même au Kurdistan irakien, les terribles stigmates de ces crimes sur les populations civiles et après aussi avoir accueilli nombre d'entre eux en France avec des associations comme la credo ou l'Oeuvre d'Orient, j'avais redemander à notre ministre des Affaires étrangères de plaider pour que le le Conseil de sécurité de l'ONU saisisse la Cour pénale internationale, il m'a répondu, ici même, que la France avait un rôle d'encouragement aujourd'hui grâce au texte, Bruno Retailleau, nous pouvons enfin aller plus loin, nous pouvons agir